Monsieur le président,

La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.-

Je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement de votre engagement tout au long de nos échanges. Ils ont été respectueux, constructifs, intenses aussi, puisque, depuis la présentation du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, nous avons eu au total près de cent heures de débat avec les parlementaires. Au terme de ce long cheminement de la rue de l'Université à celle de Vaugirard, je ne doute pas que vous connaissiez toutes et tous ce projet de loi à la lettre. Je me contenterai donc d'en rappeler l'esprit. loi comprend deux volets : le premier porte sur la confiance et concrétise l'engagement du Président de la République d'un droit à l'erreur pour les particuliers comme pour les entreprises ; le second concerne la simplification des démarches administratives. Ce projet de loi est l'un des deux piliers d'un cadre équilibré en matière de relations entre l'administration et ses usagers. Le premier pilier, dont nous allons continuer de débattre ensemble, est celui de la bienveillance vis-à-vis de l'usager de bonne foi. Le second, que Gérald Darmanin défend aujourd'hui même devant votre assemblée et devant l'Assemblée nationale, est le renforcement de notre politique de lutte contre la fraude. Contre tous ceux qui enfreignent volontairement les règles, l'État ne doit faire preuve d'aucune faiblesse ni d'aucune tolérance.

Je pense notamment à l'encadrement de la durée de contrôle par l'URSSAF pour les entreprises de moins de vingt salariés ou à l'extension du rôle des commissions des impôts directs et des taxes, au sein desquelles siègent des professionnels. Le Gouvernement souhaite que cette nouvelle lecture se déroule dans l'exact même état d'esprit. Nous ferons ainsi preuve de la même écoute. Nous continuerons aussi à respecter deux principes qui nous paraissent essentiels.

On en parle peu, mais c'est là un changement concret dans le fonctionnement de nos administrations. Par ailleurs, nous oeuvrons aussi pour diminuer de manière extrêmement sévère le nombre de circulaires et, surtout, pour supprimer celles qui sont devenues obsolètes. Deuxièmement, le projet de loi porte sur la seule relation entre l'administration et les usagers. Cela continue, je le sais, d'être un motif de désaccord entre la majorité sénatoriale et le Gouvernement. Nous considérons qu'il n'a pas vocation à régler les relations entre les différentes administrations, notamment entre l'État et les collectivités territoriales. À l'inverse, grâce, notamment, à votre vigilance, nous avons tenu à ce que l'ensemble des propositions nées des débats n'induisent pas de charges ou de complexité supplémentaires pour les collectivités territoriales. C'est d'autant plus justifié alors que nous avons engagé avec elles une politique de contractualisation. Le temps législatif est, certes, essentiel ; en même temps, le rendez-vous que nous ne devons pas manquer est celui de l'exécution. Nous avons déjà commencé à nous y atteler, car, en matière d'action publique, il n'y a que les preuves qui comptent. L'ensemble des décrets d'application seront publiés avant le 31 décembre 2018.

disposition. La mise en oeuvre opérationnelle du texte est aussi à privilégier. Ainsi, nous allons accompagner de façon inédite la mise en oeuvre effective de la loi. Outre les initiatives déjà lancées sur lesquelles nous allons nous appuyer, comme l'élargissement des horaires des services publics, nous allons construire avec les usagers et les agents les modalités concrètes de mise en oeuvre des dispositions du texte, en mobilisant toutes les forces vives dans les territoires pilotes. À partir de ces territoires, nous pourrons tirer tous les enseignements nécessaires à la mise en oeuvre effective de la loi dans tout le pays. dans tout le pays. Ainsi, le référent unique pour les entreprises sera expérimenté dans le Pas-de-Calais, en Côte-d'Or et dans le Maine-et-Loire, en repartant des besoins des entreprises et des dynamiques locales existantes. Nous fonctionnerons ainsi pour tous les grands chantiers de la future loi. Les administrations sont d'ores et déjà à la tâche, afin de lancer ces travaux sitôt la loi promulguée. Par ailleurs, pour maintenir une pression- bienveillante, évidemment -sur l'exécution de la loi, nous aurons besoin de l'ensemble des parlementaires, besoin de vous toutes et tous. par l'exercice de vos missions d'évaluation traditionnelles, mais aussi par le Conseil de la réforme porté par les députés et auquel nous souhaitons que des sénateurs puissent être associés. Nous apporterons tout notre appui à cette initiative en mobilisant nos administrations. la loi seule, votée, exécutée et suivie par nous tous, ne suffira pas. Nous sommes conscients que nous aurons besoin d'investir. Tel est le sens des annonces faites le 20 juin dernier avec Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État, en ce qui concerne les lauréats du Fonds pour la transformation de l'action publique.

Ce fonds inscrit pleinement ses investissements dans le cadre de la nouvelle société de confiance. De même, quand une procédure est dématérialisée, notre seule volonté est de simplifier la vie des usagers, celle des administrations et de réduire le risque d'erreur. Ce même effort d'investissement, nous le ferons pour la formation des agents publics. C'est l'une des actions prioritaires du schéma directeur 2018-2020 pour la formation professionnelle des agents de l'État, qui vise à diffuser auprès de l'ensemble des agents une culture renouvelée de la relation à l'usager, fondée sur l'accompagnement, le conseil et la bienveillance. Pour la seule année 2018, 250 millions d'euros de crédits de formation ont d'ores et déjà été réorientés autour des objectifs de transformation de l'action publique. Enfin, pour mesurer les effets concrets de ces transformations, nous ferons preuve de transparence vis-à-vis de l'ensemble des Français. Nous suivrons l'évolution de leurs relations avec l'administration et la progression de la confiance par la mise en place d'un baromètre de la confiance, dont nous rendrons les résultats publics chaque année.

de loi avait suscité beaucoup d'attentes avant même son dépôt. Malgré une certaine déception quant à son véritable contenu, nous avions choisi d'aborder son examen de manière constructive. À cet esprit d'ouverture du Sénat, les députés de la majorité ont opposé une fin de non-recevoir, leur intransigeance conduisant à l'échec de la Quel mépris à l'égard du travail accompli par le Sénat pour enrichir et clarifier le texte initial ! Malgré tout, nous continuons à rechercher le compromis, et une convergence demeure possible. S'agissant de l'article 2, qui crée un droit à l'erreur et un droit au contrôle au bénéfice des usagers dans leurs relations avec l'administration, l'Assemblée nationale a rétabli le texte issu de ses travaux en première lecture, sans vraiment examiner le travail du Sénat. Notre commission spéciale a donc rétabli le texte du Sénat, qui ne visait qu'à préciser et à rendre plus incitatif le dispositif proposé. L'Assemblée nationale a supprimé l'extension du droit à l'erreur aux collectivités territoriales dans leurs relations avec l'État. Or je demeure convaincue de son utilité, comme vous, je pense, mes chers collègues. J'ai donc proposé à la commission spéciale, qui l'a adoptée, une rédaction de compromis réservant le bénéfice du dispositif aux plus petites communes et aux EPCI les plus modestes. De nombreux maires nous font part régulièrement de leurs difficultés d'interprétation des textes. Ce droit à l'erreur doit leur apporter davantage de sécurité juridique. Je comprends la volonté de certains d'entre vous de ne pas opérer de distinction entre collectivités et d'ouvrir le dispositif plus largement. plus largement. Je m'en remettrai à la sagesse de notre assemblée sur ce sujet. Par ailleurs, je pense que nous pouvons nous féliciter de l'adoption par l'Assemblée nationale du report de trois ans, au 1 juillet 2021, de l'inclusion des élus locaux et des fonctionnaires dans le champ d'application du répertoire numérique des représentations d'intérêts prévu par la loi Sapin II. Cette avancée est à mettre au crédit du Sénat. Si la commission mixte paritaire n'a pas abouti, ce n'est pas, en tout cas, à cause des dispositions fiscales du projet de loi. Tout d'abord, plusieurs dispositions ont fait l'objet d'une adoption conforme en première lecture, dont la garantie fiscale, l'une des avancées les plus notables du texte en faveur des contribuables. Dans le même esprit, le Sénat avait introduit un article additionnel prévoyant que, à l'issue d'un contrôle, le courrier adressé au contribuable mentionnerait non seulement les points faisant l'objet de rectifications, mais aussi les points que le vérificateur a examinés et qu'il considère comme conformes à la loi fiscale. Les députés ont apporté leur soutien à cette mesure et l'ont étendue aux contributions indirectes. Introduite par le Sénat, la dispense d'obligation de télédéclaration pour les contribuables résidant dans une zone blanche a été maintenue par l'Assemblée nationale. définitive, rien d'ambitieux dans ce projet de loi. Le droit à l'erreur existe en effet depuis bien longtemps en matière fiscale. Trois motifs importants de désaccord demeurent sur les articles fiscaux du projet de loi, mais nous ne perdons pas espoir d'aboutir à un compromis. Premièrement, l'article prévoyant la publication des rescrits, que l'Assemblée nationale a supprimé, a été rétabli par notre commission spéciale dans une rédaction de compromis, limitée aux demandes présentant un intérêt général, et non plus une portée générale, de façon à laisser une plus grande marge d'appréciation à l'administration. Deuxièmement, en ce qui concerne l'ouverture au public des données relatives aux transactions immobilières, nous avons choisi de rétablir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée, mais dans une version de compromis compatible avec un dispositif d'.

confiance, tout en conservant un apport bienvenu des députés, qui permettrait à l'administration de labelliser les sociétés engagées dans le dispositif dans une logique de responsabilité fiscale des entreprises. J'en viens aux dispositions touchant aux affaires sociales. En ce qui concerne la médiation, l'Assemblée nationale a créé un dispositif juridique commun à l'ensemble des branches du régime général de la sécurité sociale, tenant compte de nos préoccupations. de loi prévoit aussi, à titre expérimental, un cadre dérogatoire au droit du travail pour permettre la mise en place de prestations de relayage des proches aidants. Nous rétablirons l'encadrement de cette expérimentation, en rendant applicable la convention collective des salariés du particulier employeur. De même, nous rétablirons un article modulant le montant de l'annulation des exonérations de cotisations sociales encourue par l'employeur lorsqu'il omet de déclarer certaines heures supplémentaires ou qu'une prestation de services est requalifiée en travail salarié. Enfin, je vous proposerai à nouveau de supprimer l'habilitation demandée par le Gouvernement pour réformer par ordonnances les règles qui régissent les modes d'accueil du jeune enfant. Outre qu'il s'agit clairement d'un cavalier législatif,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en première lecture, le Sénat avait cherché à donner plus de substance à ce projet de loi un peu fourre-tout. Malgré notre volonté d'aboutir, la commission mixte paritaire a échoué sur deux points, dont l'un, portant sur les éoliennes en mer, n'avait été voté ni par l'Assemblée nationale ni par le Sénat, ce qui est tout de même assez inédit. Pour cette nouvelle lecture, nous avons à nouveau choisi de jouer le jeu en améliorant le texte, car nous ne désespérons pas que le Gouvernement ou nos collègues députés finissent par nous entendre. En matière de rescrit, l'Assemblée nationale a certes conservé les procédures sectorielles introduites par le Sénat, mais elle les a complétées de nombreux dispositifs inédits dans des domaines variés au mépris de la règle de l'entonnoir. Notre commission les a donc supprimés. S'agissant du rescrit en matière juridictionnelle, nous avons adopté une solution de compromis qui permet de conserver le dispositif du Gouvernement tout en précisant son champ d'application. L'expérimentation sera limitée aux décisions relatives aux déclarations d'utilité publique et aux déclarations d'insalubrité, ce qui évitera d'engorger les juridictions administratives. En matière d'information des usagers, notre commission a de nouveau ramené le délai maximal de délivrance du certificat d'information à trois mois, ce qui suffira amplement puisqu'il s'agit simplement de lister les règles applicables à une activité et non de les interpréter. Concernant la désignation de référents unique dans les maisons de service au public, malgré nos réticences sur le principe, nous avons également adopté une rédaction de compromis qui permettra de s'assurer de l'accord de tous les participants. La commission a en revanche rétabli la modulation de la durée des contrôles administratifs que nous avions introduite en première lecture au profit des TPE. Cette différenciation est à la fois légitime sur le fond et parfaitement réalisable sur le plan pratique. De même, nous sommes également revenus à notre texte afin de garantir que les transferts de compétences des chambres départementales d'agriculture aux chambres régionales ne puissent être expérimentés qu'avec l'accord des intéressées, car nous croyons en la capacité des acteurs territoriaux à s'organiser de la façon la plus efficace possible sans qu'il faille les y contraindre. En matière d'enseignement supérieur, je me réjouis que les députés aient confirmé le délai d'habilitation fixé à six mois par le Sénat et que les modalités de sortie de l'expérimentation des regroupements aient été sécurisées. Concernant la participation du public aux projets qui ont une incidence sur l'environnement, l'Assemblée nationale a rétabli la possibilité de remplacer l'enquête publique par une consultation par voie électronique. Elle est même allée plus loin que le texte initial, qui limitait cette expérimentation aux seuls projets agricoles, en l'étendant à l'ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, c'est-à-dire à tous les projets d'installations classées. Considérant que l'enquête publique est nécessaire pour permettre l'acceptabilité des projets, nous avons de nouveau supprimé cette expérimentation. Le Gouvernement a aussi profité de la nouvelle lecture pour faire ratifier l'ordonnance de 2017 sur l'autorisation environnementale. Une telle ratification par voie d'amendement porte atteinte aux droits du Parlement, qui ne dispose pas du temps nécessaire pour examiner le texte et y apporter si besoin des modifications. C'est pourquoi nous l'avons supprimée. S'agissant des éoliennes en mer, chacun a en tête l'émoi suscité par l'amendement qu'avait présenté le Gouvernement pour renégocier sous la menace d'une annulation le prix des six parcs déjà attribués et notre opposition quasi unanime en première lecture.

Malgré ce résultat favorable, la façon dont le Gouvernement a géré ce dossier doit nous interpeller. Sur le fond, si l'amendement a certainement joué comme un levier dans les négociations, pourquoi le maintenir malgré l'aboutissement En droit, l'État pourra toujours annuler les décisions d'attribution jusqu'à la signature des contrats d'achat. Nous ne savons rien, du reste, de la manière dont l'accord a été formalisé, de ses conséquences éventuelles sur l'emploi et sur la filière industrielle ou encore de la façon dont les économies annoncées ont été calculées. Je suppose toutefois que vous nous donnerez un certain nombre d'informations sur ce sujet, J'ajoute que ces dernières ont été en partie gonflées, puisque le coût du raccordement, jusqu'alors intégré dans le tarif d'achat, sera désormais couvert par le tarif d'utilisation des réseaux : c'est près de 1,2 milliard d'euros que l'on fera ainsi passer d'une ligne de facture à l'autre. De même, l'occupation du domaine public à titre gratuit occasionnera une perte de recettes publiques de l'ordre de 360 millions d'euros qui n'est pas comptabilisée. Enfin, la possibilité pour l'État de revenir sur des accords déjà conclus est un mauvais signal envoyé aux entreprises qui souhaitent investir dans notre pays, pays, dans un texte censé faire renaître la confiance. Il faut conclure ! Malgré tout, parce que le débat a déjà eu lieu en première lecture et parce qu'il faut prendre acte des résultats des négociations, nous avons choisi de ne pas y revenir. La parole

cent trente ans jour pour jour, Wolfgang Amadeus Mozart achevait la composition de la symphonie n° 40, qui allait devenir l'une des pièces maîtresses du répertoire. Plus aride, le texte que nous examinons une dernière fois en séance publique constitue pourtant, je veux le croire, une véritable partition pour rénover les relations entre les usagers et leurs administrations. Les Français sont attachés au service public. Le baromètre Delouvrier, qui mesure la satisfaction des usagers, indique que, en 2017, 72 % des Français étaient satisfaits, soit une progression de 5 points par rapport à 2014. Dans le même temps, il n'est pas interdit d'interroger la pertinence de ces services publics, à la lumière de la révolution numérique dans nos vies et dans nos villes. M. Thierry Tuot, conseiller d'État, estime le coût de la suradministration à environ 3 points de PIB. 3 points de PIB. Demain, il s'agira de repenser avant de dépenser. Le droit à l'erreur est devenu, au gré de nos débats, la mesure phare de ce projet de loi. C'est, nous le savons tous, une attente forte de nos concitoyens et de nos entreprises. Nous avons, par l'adoption d'un amendement de notre collègue Patricia Schillinger, étendu le champ de ce droit au code de la sécurité sociale. D'autres apports importants du Sénat ont été retenus. J'en ai dénombré à peu près une trentaine ; je me suis peut-être trompé, mais je crois que cela doit nous conduire à nuancer

est bien d'améliorer la relation qu'entretient le citoyen avec l'ensemble des administrations. Cette extension interroge en droit : comment une personne morale de droit public pourrait-elle se prévaloir d'un droit à l'erreur au profit de l'État La réponse est claire : le droit de la responsabilité des personnes morales est orienté vers l'administré et il obéit à des règles spéciales. De même, doit-on étendre ce droit à l'erreur aux relations entre les collectivités elles-mêmes, au risque de créer une tutelle ? Enfin, imaginons-nous un citoyen qui pourrait se prévaloir d'une erreur d'une collectivité qui ferait elle-même usage de son droit à l'erreur envers l'État ? On atteindrait un niveau d'insécurité juridique dangereux pour les Français et pour les entreprises. Je ne suis pas contre

Ces désaccords ne doivent pas occulter les apports de ce texte, qui prévoit des changements importants : présomption de bonne foi qui pèse sur l'usager, expérimentation du référent unique dans les maisons de services au public, généralisation du rescrit, limitation de la durée des contrôles sur nos TPE ou PME. Je souhaiterais m'arrêter un instant sur le titre III, intitulé « Un dispositif d'évaluation renouvelé », qui a été en partie vidé de sa substance ; je le regrette. Nous sommes tous attachés au renforcement des pouvoirs d'évaluation des politiques publiques par le Parlement, en particulier par le Sénat. Ce n'est certes pas incompatible avec la communication de rapports relatifs au suivi de l'application des bonnes pratiques ou des expérimentations par le Gouvernement, mais il est vrai qu'un bon rapport est un rapport utile.

qui peut ne pas fonctionner, mais qui aura le mérite d'exister et d'être innovante. Cela me fait penser au mot de Jules Renard : « La porcelaine cassée dure plus que la porcelaine intacte. » Tout n'est pas parfait, contrairement à Mozart, mais nous prévoyons le nécessaire pour corriger les fausses notes. Quoi qu'il en soit, les sénateurs auront à coeur d'appuyer votre action, notamment auprès des services déconcentrés de l'État, que ce soit la DGFiP ou les DIRECCTE, dans nos territoires. Le numérique est un levier de solidarité, y compris dans les grandes villes. C'est au prix de ces adaptations que nous redonnerons confiance aux jeunes générations dans l'action publique, trop longtemps cantonnée aux moyens et pas assez tournée vers les résultats. Notre crédibilité passe par un sursaut d'efficacité que le projet de loi veut encourager, et j'espère qu'il en sera l'augure. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici donc réunis pour débattre d'un projet de loi dont le moins qu'on puisse dire est qu'il a fait l'objet lors de sa présentation d'une offensive de communication pour le moins insistante.

avec le développement des contrats de mission et autres emplois contractuels. Outre que la recette est assez ancienne, comment peut-on faire de la bonne administration, avec la sécurité juridique et la confiance qui conviennent, quand on place les acteurs de ces administrations en situation d'insécurité professionnelle ? Le projet de loi ne remet nullement en question les politiques qui, de révision générale des politiques publiques en modernisation de l'action publique, ont largement entamé la crédibilité du service public par l'abandon marqué de la présence territoriale des services déconcentrés des différentes administrations. qu'il les prolonge et en accentue les défauts et travers, pour faire de cas d'espèce la matrice de la suraccumulation législative que nous connaissons. fait ainsi cohabiter des mesures à caractère général avec des mesures tout à fait circonstanciées ou circonstancielles dont nous pouvons nous demander, au demeurant, ce qui les a inspirées. simplement la volonté de répondre aux attentes d'on ne sait quel groupe de pression ou groupement d'intérêts désireux de bénéficier de l'onction de la loi pour prolonger son action. Il est vrai que, depuis un an, nous ne sommes plus dans le régime des partis- normalement, vous devriez applaudir -, mais que nous sommes passés à celui des lobbies, du mouvementisme, de la confusion des genres pouvant aller jusqu'à la sécurité des déplacements présidentiels Sur le strict plan du droit, qui doit être le même pour tous, fondé sur l'égalité entre les citoyens, nous ne sommes pas certains, à l'instar du Défenseur des droits, que ce texte apporte beaucoup. Outre qu'il va sans doute accuser les effets de la fracture numérique, à peu près irréversible tant que vivront en France des personnes nées avant la Seconde Guerre mondiale, le projet de loi risque de voir les dispositifs envisagés bénéficier essentiellement aux personnes déjà les plus à même de les mobiliser et de renforcer ainsi les inégalités d'accès au droit- c'est n'est pas que moi qui le dis, c'est aussi M. Toubon. Il est évident que, dans la société de confiance décrite par le texte, excusez-moi cette formule, mais elle a le mérite d'être explicite, ce sera avocat-conseil pour les uns

On ne peut enfin que souligner les liens existant entre ce texte et la conception de l'entreprise que portent le Gouvernement et sa majorité. Ils se situent en effet dans le droit fil des seules attentes des conseils d'administration de groupes industriels et financiers, attentes caractérisées par le respect de normes minimales au plan social, économique, administratif ou comptable. Qu'est-ce donc, par exemple, sur le prélèvement à la source dans les entreprises de moins de vingt salariés ? D'un côté, on a une exigence croissante de l'irresponsabilité sociale et, de l'autre, une perception de ressources publiques sans cesse plus importante ! Avec ce projet de loi, il sera demain nettement plus facile de frauder l'impôt sur les sociétés que d'obtenir illicitement une allocation de RSA. Qu'est-ce donc que cette société de confiance qui va passer la main sur la fraude au petit pied et ne va pas se donner les moyens de poursuivre la grande délinquance financière ?

collègues, nous partageons la philosophie de ce texte. Nous croyons en cette société de confiance qu'appelle le projet de loi. Nous saluons les mesures de simplification qu'il porte et nous nous félicitons, entre autres dispositions, de la suppression des sanctions pour toute première erreur d'un usager de bonne foi. Nous restons cependant en alerte et pour le moins perplexes sur de nombreux points. Après l'échec de la commission mixte paritaire et le renvoi en nouvelle lecture qui nous réunit aujourd'hui, de nombreuses dispositions que nous avions votées avec la majorité sénatoriale ont été supprimées. Nous saluons le nouveau travail des rapporteurs et des sénatrices et sénateurs de la commission spéciale, notamment sur le droit à l'erreur au bénéfice des collectivités ou sur la suppression de l'article concernant les modes d'accueil de la petite enfance- disposition plutôt incongrue, les modes d'accueil de la petite enfance ne pouvant se négocier à moindre formation et à moindre encadrement. Nous saluons également les mesures en faveur des chambres d'agriculture. Cette nouvelle lecture nous donne l'occasion de revenir sur des points problématiques que j'articulerai autour de deux axes. Le premier porte sur l'esprit général du texte. Les mesures portées dans le projet de loi- nous ne le répéterons jamais assez -touchent à des domaines multiples.

Le titre I vise à créer les conditions d'une confiance retrouvée du public dans l'administration en concentrant l'action de cette dernière sur ses missions d'accueil et de conseil. Peut-on y répondre en restreignant le champ de l'accès au droit ? La confiance dans l'administration n'est pas exclusivement celle des entreprises ; elle est également celle des citoyens. À cet égard, il me semble que l'administration n'est pas aujourd'hui en mesure d'accompagner les plus fragiles. Le Défenseur des droits, que nous avons auditionné, a pointé une fracture numérique qui touche les publics vulnérables. Beaucoup trop de nos concitoyens ne bénéficient pas des droits et des services auxquels ils peuvent prétendre. Ils sont des millions ! Il est nécessaire de restaurer la confiance afin qu'elle puisse profiter à tous. Une enquête de 2017 publiée par le Défenseur des droits souligne que 27 % des Français n'ont pas accès à internet ou éprouvent des difficultés à réaliser leurs démarches administratives sur internet.

La commission a refusé d'inscrire dans la stratégie nationale cette prise en compte de la marginalisation numérique pour que les économies réalisées par la dématérialisation profitent à la réduction de cette fracture. Or, aujourd'hui, 15 % des foyers n'ont pas accès à internet, 500 communes sont considérées comme des zones blanches

Le texte que nous examinons ne nous semble pas non plus répondre à la question des moyens. L'extension du champ du rescrit, par exemple, peut-elle vraiment s'articuler avec une baisse du nombre de fonctionnaires ? En clair, plus de travail et moins de moyens Le risque est d'ores et déjà annoncé : une modification des responsabilités et des tâches des fonctionnaires. Je m'attacherai à présent à certaines mesures clés du texte. Pour commencer, je ne peux que féliciter la commission spéciale pour son travail sur l'extension du droit à régularisation en cas d'erreur au bénéfice des collectivités territoriales. Comme les usagers de l'administration, elles ont besoin du regard bienveillant de l'État dans le cadre des missions quotidiennes qu'elles effectuent. Il s'agit d'un marqueur à leur égard. Je pense tout particulièrement aux petites communes, qui sont souvent- nous ne pouvons que le regretter -démunies face à la complexité juridique des procédures dont elles ont la charge. Monsieur le secrétaire d'État, au vu des sujets entrant dans le cadre de l'examen de ce texte, et par esprit d'équité,

J'en appelle à votre vigilance quand nous examinerons cet amendement, car nos agriculteurs doivent eux aussi faire face à la complexité croissante des dossiers sans pour autant bénéficier d'un appui technique pour les remplir. L'agriculture est un secteur clé qui ne saurait être négligé dans ce projet de loi. Le doute est aussi très fort sur l'expérimentation de la régionalisation des chambres d'agriculture. Monsieur le secrétaire d'État, j'espère que le point de vue du Sénat sur l'article 19 sera entendu par l'Assemblée Le transfert aux chambres régionales d'agriculture des missions des chambres départementales ne peut en aucun cas se faire sans l'accord de ces dernières. Plus surprenant et clivant, enfin, le retrait des associations cultuelles du champ des représentants d'intérêts. La loi relative à la transparence de la vie publique, dite Sapin II, avait tranché le débat en définissant un représentant d'intérêts comme une organisation de droit privé qui exerce régulièrement une activité ayant pour finalité d'influencer la décision publique, notamment en matière législative ou réglementaire, et entrant en communication avec des décideurs publics. Notre logique n'est pas de discriminer, mais de rétablir l'obligation pour les associations religieuses de se déclarer comme telles. D'ailleurs, qui pourrait encore soutenir que les associations religieuses n'ont pas eu d'influence sur les parlementaires, et cela dans un passé très récent ? C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Un sentiment d'étonnement s'impose quand on compare votre empressement à renouer la confiance avec les associations cultuelles

Pourquoi remettre en cause l'une des valeurs fortes de notre République, la laïcité, quand ce texte en appelle à une confiance retrouvée du public avec l'administration ? Nous en appelons en toute logique à une cohérence dans la transparence de la vie publique. L'actualité m'oblige à vous faire remarquer que cette transparence et cette confiance que vous appelez, nous souhaiterions également et avant tout la voir portée au plus haut sommet de l'État. Vous l'aurez compris, sans évolution notable sur les sujets qui nous opposent, le groupe socialiste et républicain s'abstiendra sur ce texte. La parole

un texte qui peut être mis en perspective avec le discours du Président de la République devant le Congrès et avec vos annonces datant du début du mois, monsieur le secrétaire d'État, sur la réforme de vos services. Le Gouvernement souhaite faire du retour de la confiance un axe majeur de son action. Il y réussit assez bien pour nos concitoyens, pour nos entreprises et pour les investisseurs, qui ont retrouvé confiance dans l'économie française. Il y réussit moins avec les élus locaux et avec les collectivités, avec lesquels la distance est malheureusement encore la règle, même si je connais votre souci des territoires, Ce texte participe du choc de confiance que vous voulez créer à tous les niveaux de la société. Son importance tient avant tout à l'ambition d'un véritable changement de culture au sein de l'administration. Cela fait des années que nous essayons d'instaurer une culture de la confiance entre les administrations, les citoyens et les entreprises. Cela fait des années que nous cherchons à créer une administration plus responsable, plus ouverte, plus diligente et respectueuse des intérêts des forces vives de la Nation. Sans confiance, il ne peut y avoir ni sécurité juridique, ni croissance économique, ni surtout d'unité nationale. Nous déplorons ainsi l'échec de la commission mixte paritaire, mais les désaccords étaient trop profonds. La commission spéciale du Sénat, présidée par Jean-François Husson, avait pourtant pris l'initiative de nombreux amendements pragmatiques de clarification, de précision ou tout simplement de suppression des dispositions les moins pertinentes. Elle avait également permis des évolutions substantielles, comme l'extension du bénéfice du droit à l'erreur aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Nous avions toutefois regretté en première lecture que cette volonté d'efficacité et de bon sens ait été poussée un peu loin sur certaines parties du texte. De même, la chasse légitime de notre commission à l'incompétence négative avait conduit à vider de leur substance plusieurs dispositions intéressantes du texte issu de de l'Assemblée nationale. Ces changements ont paru trop importants à nos collègues députés pour être pris en compte. Reconnaissons néanmoins, monsieur le secrétaire d'État, que tout n'est pas à jeter dans ce texte du Sénat, qui a beaucoup travaillé, et de façon constructive. du droit à l'erreur des collectivités territoriales, nous espérons des réponses plus étoffées que la position de principe selon laquelle celles-ci ne sont pas des usagers. Certes, mais les petites communes se trouvent souvent dans des situations comparables à celle d'usagers fragiles face à la complexité des normes et des procédures. Vous nous proposez, dans le projet de réforme constitutionnelle, un droit à la différenciation des collectivités. Vous nous avez annoncé, monsieur le secrétaire d'État, une déconcentration de proximité de la part de l'administration fiscale. Allons au bout de la logique, et je vous le propose, admettons, sinon un droit à l'erreur des collectivités, du moins une meilleure articulation entre la décentralisation et la déconcentration dont les rythmes différents déboussolent parfois les élus et les usagers. Enfin, je voudrais conclure en rappelant les responsabilités qui pèsent sur l'administration dans la mise en oeuvre de ce texte. Celui-ci appelle en effet de nombreuses expérimentations, de nombreuses habilitations, de nombreux décrets d'application et des exigences d'évaluation. En un mot, une grande responsabilité pèse sur le Gouvernement et les administrations pour faire de ce texte une réussite concrète et tangible. L'adoption de ce texte doit être non pas une fin, mais le début d'une nouvelle logique pour l'administration. Celle-ci sera largement responsable de son échec ou de son succès. Alors que vous commencez la restructuration de vos services, c'est autour de cette nouvelle logique de conseil et d'accompagnement que les équipes et les pratiques doivent être rénovées. En fin de compte, ce texte n'est qu'un début : l'administration devra mériter, en se réformant, la confiance que le législateur et l'ensemble des Français placeront en elle pour simplifier et améliorer leur quotidien. La parole

en nouvelle lecture, le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. « L'erreur est humaine, mais l'entêtement [dans son erreur] est diabolique. » Cette formule attribuée à Sénèque- cela fera Savoldelli -garde toute sa modernité tant à l'adresse de nos collègues députés que pour ce qui concerne ce projet de loi, dont la principale mesure tend à généraliser le droit à l'erreur dans les relations entre l'administration et les administrés, particuliers comme entreprises. Cela a été dit et répété, il s'agit d'un texte attrape-tout. Si le titre I comporte bien des mesures relatives au droit à l'erreur- lors de contrôles visant les usagers en matière de prestations sociales, en l'absence de certaines pièces justificatives dans la constitution d'un dossier, par l'extension et la généralisation de la pratique du rescrit -, les titres suivants sont porteurs de mesures les plus diverses : expérimentation de simplification dans la délivrance de titres, mutualisation de gestion de certificats de pensionnés de retraite, nombreuses habilitations à légiférer par ordonnance dans le domaine de la construction, accueil de la petite enfance, régime de responsabilité des agences de notation de crédit, et j'en passe. Aussi, et afin de conserver le cap que mon groupe s'était fixé en première lecture et pour ne pas surcharger inutilement les débats en cette fin de soirée et de session extraordinaire, je concentrerai mon propos sur quelques points qui me paraissent particulièrement essentiels et qui n'ont, à mon sens, pas leur place dans ce projet de loi. Je veux d'abord parler de l'article 38 visant, notamment, à supprimer l'obligation d'inscription au registre des représentants d'intérêts pour les associations cultuelles. Si je remercie M. le secrétaire d'État Olivier Dussopt du compromis trouvé sur les revenus cultuels tirés d'immeubles de rapport, une promesse tenue promesse tenue comme à votre habitude, ... Très bien ! ... la question du registre, que nous avions déjà soulevée en première lecture, continue, quant à elle, de poser des difficultés importantes. Je regrette que nous n'ayons pu parvenir à un accord ni en commission spéciale ni avec le Gouvernement sur ce point. Si elle est adoptée en l'état, cette disposition constituera un recul important par rapport à la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il n'y a rien de choquant à ce que les associations cultuelles fassent du lobbying et qu'elles soient considérées comme des représentants d'intérêts comme les autres auprès du parlement français et des pouvoirs publics ; c'est déjà le cas au niveau européen. Comme d'autres acteurs de la société civile, ces associations peuvent intervenir dans le débat public, dans le respect de la loi de 1905 et de l'article 1 de la Constitution, mais elles doivent le faire en toute transparence.

portant habilitation à restructurer les réseaux de chambres d'agriculture par voie d'ordonnance. Malgré des améliorations apportées en commission spéciale, avec une meilleure prise en compte des prérogatives des chambres départementales, je continue à considérer que cette mesure est un cavalier législatif, préjudiciable aux réseaux de chambres d'agriculture. Enfin, avec mon collègue Franck Menonville et en complémentarité avec le groupe socialiste et républicain, nous souhaitons nous associer à la volonté de garantir le droit à l'erreur dans l'application des règles administratives de la PAC, la politique agricole commune, qui posent tant de difficultés aux agriculteurs, un droit qui n'est pas assuré par le projet de loi dans sa rédaction actuelle et qu'il faut établir. J'apporterai également mon plein soutien à l'amendement, adopté de nouveau par la commission spéciale, visant à garantir un droit à régularisation en cas d'erreur pour les collectivités territoriales. Les collectivités et leurs groupements ont effectivement besoin du regard bienveillant de l'État et des organismes de sécurité sociale dans les missions qu'ils accomplissent au quotidien et dans le cadre des procédures qu'ils engagent. Ainsi, avec cette disposition, nous aurions un dispositif complet garantissant une administration à l'écoute de tous les usagers, citoyens, entreprises et collectivités. Lors de la première lecture, la majorité des membres du RDSE se sont abstenus sur le vote de ce projet de loi. Nous conditionnons, comme en première lecture, notre vote à l'adoption des amendements précités et, plus précisément, de celui qui porte sur la suppression de l'alinéa 2 de l'article 38 et l'obligation d'inscription des associations cultuelles au registre des représentants d'intérêts que nous demandons.

nos débats dans la nuit -pour procéder à une nouvelle lecture du projet de loi dit « pour un État au service d'une société de confiance ». Il s'agit d'un texte aux ambitions multiples, dont l'objet central est de promouvoir l'établissement d'une nouvelle relation entre l'État et les citoyens, en leur qualité d'usagers de l'administration. Cette relation se veut être basée sur la confiance. Je pense que nous pouvons tous ici appeler de nos voeux l'émergence d'une telle « société de confiance », même si l'on pourrait nous opposer que, au cours des derniers mois, le Gouvernement a semblé peu disposé à suivre cette voie : non-communication du rapport du Comité Action publique 2022 aux membres dudit comité ; échec de la négociation dans la mise en oeuvre du dispositif de contractualisation avec les collectivités locales, deux exemples emblématiques parmi d'autres qui incitent plutôt à la méfiance. Instaurer cette relation de confiance nécessite d'ajuster et de moderniser la pratique administrative. Le droit à l'erreur constitue une innovation intéressante en ce qu'il écarte la possibilité de sanctionner le citoyen ayant commis une erreur de bonne foi et cherchant à la régulariser. Ce dispositif présente l'avantage de sortir l'administré de l'état de suspicion presque systématique qui prévalait jusqu'ici : après tout, si la présomption d'innocence guide notre procédure pénale, la même démarche ne serait-elle pas tout aussi naturelle dans les relations entre administration et administrés ? Le droit au contrôle, contrepartie du droit à l'erreur, ouvre un droit pour le citoyen d'être contrôlé et donc de pouvoir s'assurer qu'il respecte bien la norme. Mettre en oeuvre ces deux droits permet d'établir les conditions d'une confiance mutuelle : pour l'administration, le citoyen ne sera plus systématiquement présumé comme étant délibérément en faute, tandis que, pour ses interlocuteurs, l'administration ne sera plus vue comme disposée à systématiquement les sanctionner, y compris ceux qui le seraient de bonne foi. Autour de ce diptyque s'articulent de nombreuses autres mesures. Le rapport de certaines d'entre elles avec l'objet général du projet de loi est parfois ténu. Cela a conduit le Sénat à proposer une nouvelle dénomination de ce texte fourre-tout, « attrape-tout », multipliant les mesures expérimentales ou les habilitations à légiférer par ordonnance. Le nouveau titre « projet de loi renforçant l'efficacité de l'administration pour une relation de confiance avec le public » paraissait plus en adéquation avec le contenu réel du texte. Mais les députés ont considéré que ce titre tendait à « récuser la philosophie même du projet de loi dont l'ambition est, en changeant l'État, de susciter de nouveaux comportements sociaux ». il me semble que les dispositions hétéroclites de ce texte ne sont pas la parfaite illustration de cette ambition. En effet, dans le projet de loi adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, nous trouvons de nombreuses mesures portant sur la modernisation des pratiques administratives : il s'agit notamment du développement des rescrits administratifs et autres actes opposables, du recours aux médiateurs, de la dématérialisation ou encore de l'essor du guichet unique. d'autres mesures concernant la simplification et l'évaluation des mesures administratives, comme la possibilité d'effectuer des regroupements volontaires d'établissements dans l'enseignement supérieur, la mise en place du « relayage » au domicile dans l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie ou encore la demande de plusieurs rapports au Gouvernement. des mesures plus éloignées de l'objet principal du texte, celles qui sont relatives aux énergies renouvelables, mais aussi au régime des associations cultuelles et à la responsabilité des agents publics. Notre assemblée, notamment sur l'initiative de ses deux rapporteurs, avait réalisé un important travail d'amélioration et de mise en cohérence du texte initial. Malheureusement, et en dépit des efforts des sénateurs, les discussions en commission mixte paritaire n'ont pu donner lieu à un accord. L'une des raisons de cet échec a notamment été l'insistance de nos collègues députés du groupe La République En Marche à inscrire coûte que coûte à l'article 34 des dispositions tendant à remettre en cause les résultats des appels d'offres relatifs à la production d'électricité en mer à partir de l'énergie mécanique du vent. Comme l'a si justement rappelé le rapporteur Jean-Claude Luche, si le Sénat ne peut être en désaccord avec l'objectif poursuivi, à savoir diminuer le coût de l'électricité pour les consommateurs, il ne pouvait rester muet sur la forme : des dispositions introduites par un amendement de dernière minute du Gouvernement- encore un, échappant ainsi à l'avis du Conseil d'État et à l'étude d'impact. Si l'on en croit les déclarations du Président de la République au cap Fréhel, un accord sur la renégociation des contrats a été trouvé avec les trois consortiums lauréats. lauréats. Que de temps perdu, alors même que le calendrier législatif de ces dernières semaines a été très chargé ! Je loue ici la sagesse de la commission spéciale, qui n'a pas souhaité rouvrir le débat. ce texte présente de nombreux éléments intéressants, mais dont la portée a été affaiblie par une étude d'impact jugée insuffisante par la commission spéciale, par un manque de lisibilité et par des changements d'arbitrage du Gouvernement sur des points importants. C'est, par exemple, le cas de l'article 38 relatif au statut des cultes. Était-il indispensable de traiter cette question complexe dans ce projet de loi ? Sans doute pas ! La dernière version de cet article, adoptée par l'Assemblée nationale et acceptée par la commission spéciale, a été en grande partie vidée de son contenu. Le travail législatif effectué jusqu'à présent a permis d'améliorer le texte, et nous continuerons de le faire ce soir. À l'occasion de la nouvelle lecture, les députés ont toutefois affiché leur désir d'aboutir à un compromis. Ils ont, à cette occasion, maintenu vingt et un articles dans la rédaction issue des travaux du Sénat. C'est la même volonté qui a animé les membres de la commission spéciale ; en témoigne la limitation du droit à l'erreur des collectivités territoriales aux petites communes. Cependant, sur d'autres points, comme les multiples demandes de rapport prévues aux articles 40, 41, 42 et 46, le Sénat n'a pas abandonné sa philosophie. Le ministre de l'action et des comptes publics s'est engagé devant les députés à faire en sorte que les décrets d'application soient tous publiés avant le 31 décembre 2018. Plus rien ne s'oppose désormais à ce que le projet de loi entre en vigueur et, espérons-le, instaure cette société de confiance que nous appelons tous de nos voeux.

mixte paritaire le 5 avril dernier, nous voici aujourd'hui amenés à discuter en nouvelle lecture du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Ce texte, que l'on a pu résumer en deux mots- « confiance » et « simplification » -, a nourri de nombreux espoirs avant même son dépôt. Sont ici en jeu non seulement la confiance des citoyens envers leur administration, mais également la confiance des entreprises en l'efficacité de l'État. Sur le plan de la simplification, le projet de loi procède procède du constat suivant lequel l'imbrication des procédures entrave trop souvent le bon fonctionnement des services publics, encourageant conséquemment la défiance des particuliers comme des entreprises. Ces espoirs, il faut bien le dire, ont été largement déçus. Le projet de loi transmis par l'Assemblée nationale était parsemé de mesures superfétatoires. Nous nous sommes donc attachés à les faire disparaître en commission spéciale, puis en séance publique, contribuant ainsi à ancrer le texte dans la réalité. Le Sénat s'est ainsi montré constructif, tentant de donner à ce texte une cohérence qui lui faisait défaut. Tout en supprimant un grand nombre de rapports parfaitement inutiles, nous avions cherché à sauvegarder les prérogatives du Parlement, en limitant rigoureusement la durée des habilitations à légiférer, la loi ne pouvant et ne devant se faire en permanence sans le Parlement. Pourtant, à en croire le Gouvernement et sa majorité à l'Assemblée nationale, qui n'ont pas voulu entendre nos remarques, cette attitude constructive était vaine. Ainsi, malgré notre volonté de trouver un compromis, les députés ont choisi de faire échouer la réunion de la commission mixte paritaire, butant en particulier sur la reconnaissance du droit à l'erreur au bénéfice des collectivités locales et sur la question de l'éolien en mer. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des arguments avancés en CMP. Je profite toutefois de l'occasion pour saluer la sagacité et la ténacité de la commission spéciale du Sénat et de ses rapporteurs qui, dans un esprit toujours positif et prospectif, n'ont déposé que vingt-quatre amendements. Cela prouve la volonté du Sénat de trouver un compromis, malgré les soixante-huit articles restant encore en discussion. Après ces remarques sur la forme, j'en viens maintenant au fond. Là encore, plusieurs points sont à déplorer, à commencer par l'article 2 relatif aux droits à l'erreur et au droit La commission spéciale du Sénat avait proposé plusieurs améliorations du dispositif, afin de le rendre plus incitatif, mais nous n'avons pas été écoutés par l'Assemblée nationale. C'est donc une bonne chose que la commission spéciale, par la voie d'amendements de son corapporteur, persiste à vouloir améliorer ce mécanisme. J'émets, pour ma part, plus de réserves à propos de l'article 2 A, qui prévoyait d'étendre le bénéfice du droit à l'erreur aux collectivités territoriales. Si je demeure convaincue du bien-fondé de cette disposition, je ne pense pas qu'il faille à tout prix s'engager dans des compromis et dévoyer l'esprit initial de l'article en réservant le bénéfice de cette disposition aux communes de moins de 3 500 habitants et aux EPCI dont aucune commune membre n'a plus de 3 500 habitants. Si votre proposition est compréhensible, madame la rapporteur, je ne m'en satisfais pas. Aucun seuil n'est fixé pour les administrés ou les entreprises. Aussi, parce qu'il doit en être ainsi pour les collectivités locales que nous représentons, j'ai déposé un amendement pour y remédier, comme je l'avais déjà fait en première lecture, et j'ai bien noté votre avis de sagesse bienveillante. Nous ne devons pas nous contenter de dispositions « par défaut Il est de notre devoir de ne pas stigmatiser certaines collectivités et de répondre ainsi aux attentes des maires et des exécutifs locaux. Vous l'aurez malgré tout compris, mes chers collègues, le groupe Union Centriste n'est pas opposé à l'esprit de ce texte. Les objectifs sont louables. Nous déplorons en revanche la forme du débat et le sabotage de la CMP par l'Assemblée nationale. Nous voterons bien entendu ce projet de loi, en espérant que les recommandations et améliorations du Sénat trouveront un écho auprès de nos collègues députés. Il y va de la clarté et de l'efficience des dispositifs contenus dans ce texte. Les administrations, les citoyens et les collectivités locales attendent ces mesures avec impatience : ne les décevons pas ! La parole

Il est certain que nous voulons aller plus loin encore en matière de simplification. Il est aussi certain que nous voulons réussir la mise en oeuvre de ce texte pour faire en sorte que son application soit la plus concrète possible. C'est la raison pour laquelle,

Tout d'abord, je formulerai des regrets à la suite de nombreux orateurs dans la discussion générale. Mon premier regret concerne la durée bien trop longue d'examen de ce texte,

Quel rapport entre l'efficacité de l'administration et la relation de confiance à établir avec les citoyens et les éoliennes maritimes ou les modes de garde de la petite enfance ? Mon troisième regret, enfin, c'est celui d'avoir vu dans nos débats deux conceptions différentes de ce que doit être la navette parlementaire et, plus généralement, le rôle du Parlement, entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Ensuite, je déplore l'impréparation des textes présentés par le Gouvernement. Cela conduit à des demandes d'habilitation formulées sans aucune idée de ce que seront les orientations retenues et également à des changements de cap en cours de navette qui nuisent à la clarté des débats. débats. Pour terminer sur une note plus optimiste, je veux souligner quelques motifs de satisfaction. Au cours de l'examen de ce texte, le Sénat a démontré sa capacité à moderniser

Nos débats ont été constructifs, riches, attentifs, et je tiens en cet instant à en remercier tous mes collègues ainsi que, bien évidemment, Mme et M. les rapporteurs. La commission spéciale, en faisant travailler des sénateurs de toutes les commissions sur des sujets qui ne sont pas abordés dans leurs commissions permanentes de rattachement, est un facteur d'ouverture et de cohésion. Si l'on prend en compte la globalité du projet de loi et la proportion très importante des articles adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, il est clair que les objectifs poursuivis, à savoir renforcer l'efficacité de l'administration et établir et conforter une relation de confiance avec le public, ont bien été partagés et soutenus ; c'est là l'essentiel.

Apprécier l'intérêt public et l'ensemble des enjeux très en amont devrait être « la » cause commune des élus qui ont un projet et de l'administration qui va instruire les différentes phases de ce projet. Dans la vraie vie, la réalité est tout autre : les élus foncent souvent tête baissée dans la phase d'opérationnalité et se heurtent à des administrations qui, au mieux, s'en tiennent strictement à la la lettre, sans comprendre les difficultés concrètes vécues par les élus, et qui, au pire, interprètent les textes et donnent parfois des avis divergents. Le tout crée un malaise palpable sur le terrain entre les élus et les fonctionnaires de l'État et induit surtout des blocages qui nuisent aux populations. Pourtant, les solutions et les pistes de travail existent pour redonner de la confiance aux trois parties prenantes : citoyens, élus et administrations. En premier lieu, le certificat de projet, qui est peu connu et donc peu utilisé. Cet instrument de sécurité juridique et de stabilisation du droit permet au préfet de département de notifier un engagement à un porteur de projet sur les différentes procédures à respecter et les délais de délivrance des autorisations. Expérimenté en 2014 dans différents départements, il a été pérennisé au moment de la création de l'autorisation environnementale unique en tant qu'étape préalable au dépôt du dossier d'autorisation. Cette mesure est en vigueur depuis le 1 mars 2017. Une autre solution pourrait être mise en place facilement connecter les administrations entre elles pour décloisonner l'instruction. Une « équipe projet » serait systématiquement constituée en amont, composée d'un pilote élu et d'un pilote pour l'administration. L'idée est de mettre autour de la table toutes les administrations qui, du coup, coup, ne pourront plus camper sur des positions figées qui se contredisent souvent. Enfin, je rappelle l'une des propositions issues de la mission d'information relative à la démocratie, que j'ai présidée en 2017 aux côtés de Philippe Bonnecarrère, rapporteur envisager, à long terme, la création d'une procédure continue de consultation du public couvrant toutes les phases du projet d'infrastructure et placée sous l'égide d'un garant désigné par la Commission nationale du débat public. Tout cela ne pourra se faire qu'en changeant de méthode changer la méthode de travail en passant d'un travail individuel à un travail collectif ; changer les postures et les mentalités. Comme le veut le projet de loi, l'administration doit revenir à sa source : le conseil et l'accompagnement. Monsieur Cabanel ... Pour ce faire, les équipes doivent avoir une nouvelle doctrine commune. La volonté du Gouvernement de supprimer 120 000 fonctionnaires est contradictoire avec ce désir de changement. Permettez-moi de douter de la réussite de ce projet de loi. Si vous diminuez les effectifs, cela aura pour conséquence de creuser encore le fossé entre les administrations, les citoyens et les élus.

La dématérialisation des procédures par les services publics conduit à l'exclusion d'un certain nombre d'usagers, qui se retrouvent dans l'incapacité d'accomplir leurs démarches. C'est le cas des personnes qui résident dans les zones blanches, des personnes qui ne sont pas pourvues de matériel informatique ou encore de celles qui ne maîtrisent pas l'outil numérique. Dans le même temps, le ministre de l'économie et des finances annonce une économie de plus de 60 millions d'euros grâce à la dématérialisation des feuilles d'impôts, des passeports ou des permis de conduire. Il serait souhaitable qu'une partie des gains réalisés grâce à cette dématérialisation des services publics soit consacrée au financement des services d'accueil du public, aux personnes les plus vulnérables notamment, par exemple dans les maisons de services au public. Il est important de conserver une voie alternative aux services numériques pour ne pas favoriser un processus de marginalisation numérique. C'est un fait : nous avons et garderons pour des années encore des citoyens vulnérables face au numérique. Ne les laissons pas au bord du chemin et choisissons de les accompagner

est à M. Pierre Ouzoulias. Par les hasards de l'existence, certains articles prennent un relief particulier à la lumière d'événements récents, dont je ne parlerai pas, je vous rassure, même si tout le monde comprend à quelle situation je veux faire allusion. C'est le cas de l'article une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation [ ...] ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction ». Quand on prend la liste des

j'ai présenté une série d'ajustements, adoptés par le Sénat en première lecture, et destinés à rendre le dispositif plus précis et plus incitatif, tout en renforçant l'accès à ce nouveau droit pour tous les usagers.

Parmi ces propositions, et s'agissant du droit à l'erreur, nous avons notamment adopté une définition de la fraude applicable au droit à l'erreur, qui complète celle de la mauvaise foi. Je rappelle également que le champ d'application retenu est celui des procédures dans lesquelles l'administration peut appliquer une sanction pécuniaire ou une sanction consistant dans la privation ou la suspension d'une prestation due. Ce champ est donc assez limité et concerne bien les bénéficiaires des prestations sociales.

présenter l'amendement n° 9 rectifié. Le présent projet de loi exclut de l'application du droit à l'erreur les règles issues du droit européen. Or, dans le cas de la politique agricole commune, la PAC, il existe plusieurs volets définis par les États membres. Chaque année, pour bénéficier des aides financières européennes de la PAC, les agriculteurs doivent remplir des dossiers de demande, rédigés par l'administration et les services français, dans lesquels il n'est pas rare de se perdre. Les nouveaux dispositifs de la PAC impliquent des dossiers de plus en plus complexes, et les formulaires demandent un haut degré de précision. Le travail quotidien de nos agriculteurs est rude, prenant, vous le savez. Ils n'ont aujourd'hui ni forcément le temps ni l'appui technique pour remplir ces dossiers.

loi le fait que les sanctions prises en application de la déclinaison de la politique agricole commune, laissées à l'appréciation des États membres, sont bien incluses dans le champ d'application du droit à l'erreur, puisque c'est déjà le cas. En effet, en application des dispositions qui figurent à l'article 2, chaque fois que les États membres disposeront d'une marge d'appréciation dans le prononcé d'une sanction, les agriculteurs pourront faire jouer leur droit à l'erreur dans les conditions de droit commun définies aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration, nouvellement créés par le projet de loi. En revanche, les sanctions qui doivent être prises en application du droit de l'Union européenne et qui ne sont pas laissées à l'appréciation des États membres devront être appliquées sans qu'il soit possible d'y déroger, comme le prévoient également les dispositions de l'article 2, conformément à nos engagements juridiques européens. En outre, ces amendements ont pour objet de réaffirmer ce principe pour une seule matière,

Pour les agriculteurs, c'est donc seulement lorsque l'État membre n'a pas d'autre choix que d'infliger une sanction au titre de la politique agricole commune que le droit à l'erreur ne s'appliquera pas. En revanche, chaque fois que les États membres

Si « le Gouvernement entend ainsi privilégier le dialogue et le conseil au détriment du contrôle et de la sanction et renforcer la sécurité juridique des personnes », le Conseil d'État « estime qu'en créant une procédure supplémentaire sans simplifier les normes et les procédures existantes, le mécanisme du " droit au contrôle " [ ...] n'y répond que très imparfaitement ce dispositif, dont le champ d'application est extrêmement vaste, pourrait porter atteinte au bon fonctionnement de l'administration dès lors qu'il prévoit que celle-ci est tenue de faire droit à cette demande dans un délai raisonnable sans tenir suffisamment compte de ses moyens et de ses effectifs Il « relève que les moyens des services de l'État ont souvent été fortement réduits et ne lui permettent pas toujours d'assumer ses missions premières, au risque d'exposer la responsabilité de l'État et la responsabilité pénale de ses agents

avec ses équipes de vérificateurs. Je vous invite, mes chers collègues, à vous reporter au document d'évaluation des voies et moyens, en annexe du projet de loi de finances, et notamment à la partie consacrée aux résultats du contrôle fiscal.

ce qui peut représenter beaucoup, mais concerne moins de 200 % des articles. Le contrôle sur place n'est pas fait pour le contribuable, disons « ordinaire ». On peut même penser, comme le fait le Conseil d'État, que « le projet du Gouvernement pourrait emporter des effets d'aubaine au bénéfice des personnes les plus à même de connaître le droit qui leur est applicable et de disposer, en interne, de compétences et de conseils juridiques adaptés à leur situation ». Devons-nous mettre en question l'efficacité des services chargés du contrôle fiscal, élément crucial de la lutte contre la fraude,

Le présent amendement vise à supprimer le droit au contrôle au bénéfice des usagers, prévu à l'article 2- et auquel nous tenons beaucoup -, au motif que le dispositif proposé ne tiendrait pas compte des moyens et des effectifs de l'administration. Or l'article L. 124-1 du code des relations entre le public et l'administration, nouvellement créé, prévoit bien que l'administration pourra toujours refuser de procéder à ce contrôle de manière discrétionnaire. Ce refus est possible dans plusieurs hypothèses : la demande est faite de mauvaise foi- de mauvaise foi- vous avez parlé de ces entreprises qui pourraient tenter d'agir de manière incorrecte ou abusive -ou a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

dit, le présent projet de loi n'est pas un texte de simplification, et on peut le regretter. Même si nous ne sommes pas opposés au droit au contrôle- c'est pourquoi nous nous abstiendrons sur l'amendement de notre collègue Savoldelli

lieu à un allégement des contrôles, mais à un assouplissement des motifs de recouvrement, ce qui impliquera un travail important des services de Bercy. S'agissant du droit au contrôle,

aux collectivités territoriales, notamment dans leurs rapports avec l'État et ses services, sans distinction de taille. Il s'agit de rétablir un article tel qu'il avait été adopté ici même en première lecture. projet de loi accorde le droit à l'erreur aux particuliers, aux entreprises, sans distinction de revenus ou de taille. Les collectivités territoriales ne sont pas des administrations. Ne faisons pas l'amalgame ! Elles ont des relations avec les administrations

Leur accorder le droit à l'erreur, quelle que soit leur taille, c'est donc plus que montrer de la bienveillance, c'est une marque de partenariat, donc de confiance, cette confiance que vous cherchez à obtenir, cette confiance que chacun ici juge indispensable. Quel

ce que la chambre des territoires, qui connaît bien les collectivités territoriales, a pu dire. Pour autant, je suis sûre que vous, qui connaissez également ces collectivités, saurez peut-être leur faire entendre raison cette fois-ci. Il est important

à une question écrite qui attend une réponse depuis cinq mois, ce qui semble montrer que le problème est compliqué. « La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a introduit [un article] qui prévoit l'assujettissement des seules indemnités de fonction des élus aux cotisations de sécurité sociale dès lors que ces dernières dépassent la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale. » On comprend là qu'il s'agit de collectivités d'une certaine taille. Quelques agences de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales- URSSAF -, se fondant [sur un autre article] du code de la sécurité sociale, imposent aux collectivités d'intégrer les contributions patronales de retraite supplémentaire FONPEL et CAREL à l'assiette de cotisations de sécurité sociale.

engendre des redressements de la part des URSSAF, des recours gracieux, voire des contentieux devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale. » Voilà un exemple parmi tant d'autres qui montre que le droit à l'erreur des collectivités existe, quelle que soit leur taille. Très bien ! La parole est à Mme Angèle Préville, pour explication de vote.

-disposer d'un droit à l'erreur vis-à-vis de l'État ? Qui pourrait croire qu'elle est moins bien lotie que l'État pour répondre à un certain nombre de choses ? Mais, vous avez raison, la question se pose de façon différente dans un

La mise en place de la retenue à la source poserait de tels problèmes administratifs insurmontables pour les TPE et PME qu'il s'agirait, à travers cet article, de leur laisser quelque latitude dans l'application du nouveau principe fiscal

De même, il est sans doute dommageable pour la transparence que le projet de loi PACTE entende faire un sort aux commissaires aux comptes, dispensant un certain nombre d'entreprises de s'en procurer un, au risque de ne plus disposer d'une image fidèle de la situation de l'entreprise. À la vérité, on doit quand même se demander ce que signifie cet article qui, en cas d'erreur de l'entreprise « collectrice », va faire porter la faute sur le contribuable, ce qui est tout de même un comble.

supprimer 20 000 emplois au sein de la direction générale des finances publiques ? Les moyens humains, notamment au plus près du monde réel de la base fiscale, seront sérieusement entamés.

L'article L. 49 du livre des procédures fiscales dispose : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter

En outre, ses attendus sont largement couverts, s'agissant des entreprises, par la partie réglementaire du code de commerce, portant notamment sur les centres de formalités existant dans les chambres consulaires. Ainsi, l'article D. 711-10 du code de commerce l'article D. 711-10 du code de commerce dispose : « Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription. « Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement. créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique. » En clair, le chef d'entreprise qui ne passe pas par la case « chambre de commerce » se trouve dépourvu de bien des informations promises

Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux, la chambre départementale d'agriculture élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes.

: La parole est à M. Pascal Savoldelli. Cet article prévoit une extension du champ d'investigation des commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en leur permettant de donner un avis sur les majorations de droits découlant de l'article 1729 du code général des impôts et de la qualification de certaines dépenses de travaux.

sont composées de deux représentants de l'administration fiscale, d'un expert-comptable, de deux représentants des organismes consulaires, le tout sous la présidence du président du tribunal administratif. donc de reposer une question claire : en quoi l'extension de compétences de ces commissions, dont la représentativité et la composition sont tout de même limitées, apporte-t-elle un vrai « plus » aux droits des administrés ? Nous pensons même que cela peut confiner à une forme de mélange des genres qui ne semble pas souhaitable. Un chef d'entreprise désigné par un organisme consulaire pour siéger à la commission pourrait avoir connaissance de la situation de l'un de ses concurrents, avec tout ce que cela implique en termes de confidentialité.

les problèmes posés. Je rappelle que l'administration traite près de 1,2 million de procédures de recours gracieux et près de 3 millions de procédures en contentieux, consistent le plus souvent en un échange d'informations destiné à faciliter la fixation de l'imposition. Le texte de l'article a d'ores et déjà été allégé,

la commission spéciale ? Cet amendement tend à supprimer l'article 15, qui prévoit une expérimentation du référent unique doté de pouvoirs de décision dans les maisons de services au public. Le Sénat avait supprimé cet article en première lecture, eu égard aux nombreuses difficultés de mise en oeuvre pour les collectivités territoriales- le groupe La Poste nous avait notamment fait remonter un certain nombre de remarques. Nos collègues députés ont rétabli sa rédaction en nouvelle lecture, sans prendre en compte notre mise en garde. La commission spéciale a adopté une rédaction de compromis permettant de s'assurer de l'accord de tous les participants,

de l'offre de services dans ces lieux, de manière à ce que la qualité soit systématiquement au rendez-vous. Enfin, troisièmement, vous avez évoqué, monsieur le sénateur, l'administration territoriale de l'État. Il se trouve qu'une circulaire a été adressée ce jour

qui doit pouvoir contrôler quand elle le souhaite les entreprises de son ressort territorial, en vertu de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. En effet, ces contrôles visent à garantir le respect d'un certain nombre de règles de droit en matière sociale, dans l'intérêt des salariés comme dans celui des dirigeants. Ils n'ont pas uniquement une vocation punitive

pour garantir de bonnes conditions de travail pour les salariés, vérifier la légalité des contrats de travail et contrôler la conformité des installations avec la loi. C'est pourquoi il convient d'exclure l'administration du travail, au sens de la convention n° 150 de l'OIT, du champ de la présente expérimentation.

16 , qui traite des mesures relatives au contrôle fiscal, prévoit une limitation de la durée des contrôles de l'URSSAF, notamment lorsque l'entreprise contrôlée est en difficulté au regard des normes élémentaires du droit du travail.

nous souhaitons poursuivre dans cette voie jusqu'au bout. C'est pourquoi nous avons rétabli notre rédaction, qui exige notamment l'accord des chambres départementales pour le lancement d'une expérimentation relative au transfert de compétences et de personnels, tout en acceptant l'ajout de l'Assemblée nationale, qui érige au niveau législatif des dispositions réglementaires annulées par le Conseil d'État. Nous avions voté cet article

Quel est l'avis du Gouvernement ?

établis hors de France pose de nombreux problèmes, en raison notamment d'un acheminement postal compliqué, souvent peu fiable. Ces difficultés retardent,

La multiplicité des caisses de retraite impose à ces citoyens d'effectuer plusieurs fois la même démarche, ce qui accroît les risques de retard. Dans le droit en vigueur, les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la peuvent mutualiser la gestion des certificats d'existence. D'après les témoignages recueillis, elles ne le font pourtant pas. Cet amendement vise donc à rendre obligatoire la mutualisation de la gestion des certificats d'existence, afin de favoriser le partage des informations sur l'existence d'une personne entre toutes les caisses de retraite. Cela éviterait aux Français établis de France d'avoir à produire autant de certificats d'existence que de caisses de retraite

J'ai pu vérifier auprès des services compétents qu'une mutualisation de la gestion des certificats d'existence demandés aux pensionnés de l'étranger est en cours, sous la direction de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il est bientôt minuit. Je vous propose d'ouvrir la nuit et de prolonger notre séance afin d'achever l'examen de ce texte,

Cette mesure vise à faire bénéficier les associations cultuelles d'avantages pour compenser la diminution de leurs ressources. Or, outre que cela remet en cause la stricte séparation des églises et de l'État, l'étude d'impact ne fournit pas d'évaluation des retombées financières futures. cette disposition n'a pas sa place dans ce projet de loi, qui devrait se borner à traiter des relations entre l'administration et le public. À l'Assemblée nationale, le rapporteur a lui-même concédé l'absence de lien direct avec le texte, mais

Même avis, pour les mêmes raisons

au statut de grand établissement, sur le modèle de l'université de Lorraine, qui constitue un exemple en la matière. Cette proposition est en adéquation avec l'article 28 et l'amendement déposé par le Gouvernement en commission lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Elle répond aussi aux préconisations faites par la Cour des comptes dans son référé en date du 15 mars 2018. Sa recommandation est assez claire : «élargir la possibilité de recours à la formule du grand établissement pour abriter les regroupements d'établissements

à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur. Cet amendement vise à créer un troisième cas

D'abord, elle repose toujours sur l'inquiétude suscitée par le caractère expérimental du dispositif de l'article 28. Le Gouvernement y a répondu à l'Assemblée nationale, en permettant aux établissements créés sur le fondement de cette expérimentation d'être pérennisés avant son échéance. Ensuite, il me semble qu'elle priverait de tout effet utile l'expérimentation prévue à l'article 28 et risquerait d'inciter les établissements à adopter le statut de grand établissement, alors même que celui-ci ne serait pas forcément le plus adapté, simplement parce que la disposition ne revêtirait pas de caractère expérimental. Enfin, l'objet de l'amendement repose sur des justifications contestables. La Cour des comptes a bien recommandé d'élargir la possibilité de recourir à la formule du grand établissement, ce qui est effectivement souhaitable. Néanmoins, dans sa réponse, le Gouvernement a indiqué qu'il partageait la recommandation de la Cour et que, précisément, il entendait y répondre à travers cette expérimentation. Pour toutes ces raisons, il paraît plus prudent et raisonnable

et de la dépendance. L'expérimentation proposée permettra de déroger aux dispositions du code du travail relatives aux régimes d'équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit, à la durée minimale de repos quotidien, ainsi qu'aux stipulations

du régime d'autorisation unique ou non, sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun du plein contentieux, dans la mesure où le délai de recours des tiers est de quatre mois, contre deux mois dans le droit commun. Ce délai de quatre mois crée, spécifiquement pour l'élevage, une insécurité juridique et financière pour les exploitants. Cet amendement vise donc à aligner le délai de recours des tiers sur le délai de droit commun. Par ailleurs, les personnes ayant un intérêt à agir contre les autorisations environnementales sont informées de l'existence du projet, ainsi que de ses modalités, par les différentes procédures de consultation du public et d'évaluation environnementale que doivent respecter les projets concernés.

Cet article tend à réduire de quatre mois à deux mois les délais de recours contre les décisions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE, par exemple les autorisations d'installation.

Il m'apparaît en effet que cet article ne représente pas un point dur pour le Sénat, contrairement aux autres articles que nous avons rétablis en commission, par exemple l'article 35 , relatif à la lutte contre les recours abusifs. La commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement.

2, qui vise à supprimer l'obligation faite aux associations cultuelles de s'inscrire sur le répertoire numérique des représentants d'intérêts pour leurs relations avec les responsables publics, à l'exception des relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes. Comme c'est le cas au Parlement européen, les associations à objet cultuel sont considérées en France comme des représentants d'intérêts : elles ont « pour activité régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire En effet, les associations cultuelles sollicitent régulièrement les administrations publiques, les ministres et les parlementaires pour les sensibiliser à leur opinion et pour influer sur la prise de décision, notamment sur des questions de politique familiale, de bioéthique et de fin de vie. L'obligation instaurée par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique représente donc un progrès évident vers une plus grande transparence dans les relations entre représentants d'intérêts et décideurs publics, sans remettre en cause pour autant le principe de laïcité, la liberté de conscience et la neutralité de l'État face aux cultes., sa suppression représenterait un véritable retour en arrière, à à l'heure où l'État et l'ensemble des responsables publics se doivent de veiller au respect des principes de la loi de 1905 et de lutter contre les dérives sectaires- je dis bien « sectaires » -et le risque terroriste. Dans la continuité de la position du RDSE exprimée en première lecture et en commission spéciale, il est de nouveau proposé de supprimer cette disposition. La parole

aurait pour effet d'amoindrir la portée du registre des représentants d'intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique créé par la loi Sapin 2. Nous demandons juste que les associations cultuelles soient traitées par la loi sur le même pied que les autres représentants d'intérêts.

sujet. Nous parlons ici d'une disposition qui a été inscrite par le Gouvernement dans son projet de loi initial et dont les termes ont été adoptés par deux fois à l'Assemblée nationale, en première et en nouvelle lectures, sans aucune modification.

une réalité : au quotidien, pour des raisons souvent très pratiques, et compte tenu de la propriété publique des églises, qui est un héritage de la loi de 1905, les élus locaux dialoguent avec les représentants d'associations cultuelles.

Ces amendements ne sont pas dirigés contre les associations cultuelles. La loi d'octobre 2013 dispose que les associations cultuelles ne sont pas représentants d'intérêts dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes.

Je suis amené à en conclure que cette modification n'a aucune place dans ce texte, à moins qu'elle ne soit le résultat d'un occulte

Le scrutin est ouvert.

Nous avons très bien compris que cet amendement était un amendement d'appel reprenant les recommandations du rapport d'information de notre collègue René Danesi, remis au nom de la commission des affaires européennes et de la délégation sénatoriale aux entreprises en juin dernier. Je ne doute pas que le Gouvernement s'inspirera des recommandations de ce rapport. Néanmoins, il me semble important que le Gouvernement soit autonome dans la rédaction de son propre rapport. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue, faute de quoi l'avis sera

nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière

de la proposition de loi relative à la mise en oeuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération (texte de la